Mais ses conséquences sur le modèle de société que nous voulons et sur l'espèce humaine tout entière sont assez vertigineuses. Cet article instaure un cadre pour les recherches en matière de cellules souches pluripotentes induites, également appelées cellules iPS, qui sont capables de se multiplier indéfiniment et de se différencier en tout type de cellules qui composent l'organisme.

celles qui portent sur la différenciation de cellules iPS en gamètes et celles qui concernent l'agrégation de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires. députés y ont ajouté les recherches visant l'insertion de ces mêmes cellules dans un embryon animal en vue de son transfert chez la femelle et de la constitution d'un embryon chimérique.

pharmacologique, pourquoi ne pas les privilégier ? préciser dans la loi que les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique n'a rien d'exclusif et n'aura pas pour conséquence d'empêcher les protocoles de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines

le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoyait la déclaration des projets à l'Agence de la biomédecine, qui, le cas échéant, pouvait s'opposer à un protocole de recherche déclaré, notamment si ce dernier méconnaissait les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre I du livre II de la première partie du code de la santé publique. Parmi ces principes figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Issues d'une découverte scientifique réalisée en 2007, ces cellules sont fabriquées en laboratoire à partir de cellules adultes reprogrammées par le biais de l'injection de gènes spécifiques. Le caractère pluripotent de ces cellules soulève des questions éthiques délicates. Je pense en particulier à des recherches qui conduiraient à différencier ces cellules en gamètes et à les agréger avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires de manière à constituer des organismes dont la structure se rapproche de celle d'un embryon ou à les insérer dans un embryon. Si de telles recherches ne sont pas encore techniquement réalisables, elles le seront vraisemblablement dans un avenir proche. Au regard des enjeux de semblables recherches- il s'agit notamment des risques liés à la création d'embryons hybrides humain-animal -, il apparaît nécessaire que l'Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches pluripotentes induites et qu'elle autorise expressément leur mise en oeuvre. oeuvre. Cet amendement vise donc à soumettre ces recherches à une autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Chasseing. Cet amendement de repli tend à renforcer le contrôle de l'Agence de la biomédecine sur la manipulation d'embryons chimériques en soumettant les protocoles de recherche, non pas à déclaration, mais à autorisation.

Cet amendement vise à soumettre à un encadrement plus strict les expérimentations dès lors qu'un transfert chez la femelle d'un embryon chimérique est envisagé, en mettant en place un régime propre d'autorisation. Cette dernière serait subordonnée à la fois aux dispositions introduites par la commission spéciale au nouvel article L. 2151-7 du code de la santé publique et aux mesures d'autorisation prévues pour les protocoles de recherche sur l'embryon humain. L'Agence de la biomédecine aura à charge de définir les délais et les seuils

l'amendement COM-199, qui vise à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux verrous. Au-delà de la recherche, le transfert chez l'animal d'embryons chimériques hybrides animal-homme n'est pas sans soulever un certain nombre d'interrogations éthiques et morales morales : on peut légitimement craindre que le patrimoine génétique de l'humanité ne soit menacé. Dans son avis n° 129, le Comité consultatif national d'éthique a notamment relevé trois principaux risques liés à la création d'embryons hybrides humain-animal. premier est de susciter de nouveaux cas d'infection ou d'infestation se transmettant naturellement des animaux à l'homme et vice-versa ; le deuxième est d'aboutir à la conception d'organismes qui, au cours de leur développement, présenteraient des caractéristiques propres à l'espèce humaine- risque de représentation humaine chez l'animal ; enfin, le troisième est d'induire, par l'injection de cellules pluripotentes humaines, des modifications chez l'animal dans le sens d'une conscience ayant des caractéristiques humaines-

a récemment permis de reconnaître la nature sensible de l'animal dans le code civil, pilier du droit français. La défense de la nature, celle de notre planète et le respect des animaux vont de concert avec les droits de l'enfant, le statut de l'embryon humain et la défense des hommes que la vie place dans une situation de fragilité, et donc avec la défense de notre humanité. Le présent amendement vise ainsi à proscrire les créations de chimères animal-humain.

donc toute possibilité de gestation, et en abaissant le taux de cellules d'origine humaine à 40 % au lieu de 50 %.

Il est possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules ne sont pas des cellules embryonnaires, mais des cellules adultes somatiques. Cette recherche, nouvelle, n'est pas interdite ; elle est soumise à déclaration à l'ABM et non pas à autorisation. La méiose naturelle est un phénomène lent et complexe. Une méiose induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le gamète devait être utilisé en fécondation. Il est donc essentiel de préciser que les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune

85 tend à soumettre l'ensemble des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites à un régime d'autorisation, ce qui est manifestement disproportionné : les cellules iPS ne soulèvent pas les mêmes enjeux éthiques que l'embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines.

vise à soumettre les recherches, sensibles sur le plan éthique, réalisées sur des cellules souches pluripotentes induites à un régime d'autorisation préalable, en lieu et place d'un régime de déclaration. Le dispositif prévu par l'article 15 présente toutefois des garanties suffisantes pour assurer le respect, au cours de ces recherches, des principes éthiques fondamentaux. L'Agence de la biomédecine peut en effet s'opposer à tout protocole violant ces principes et toute décision d'opposition sera précédée d'un avis public de son conseil d'orientation. L'avis de la commission spéciale est défavorable.

l'amendement n° 84 rectifié, la commission spéciale a précisé à l'article 14 que la création d'embryons humains par fusion de gamètes était interdite. Cette interdiction s'applique à tous les gamètes humains, mais la précision que comporte l'amendement permet de la renforcer, s'agissant de la fécondation de gamètes produits par différenciation

par cohérence avec la suppression de l'article 17 et donc du maintien de l'interdiction absolue des embryons chimériques, il convient, selon moi, de supprimer toute mention dans l'article 15 d'une possibilité de recherches conduisant à un embryon chimérique avec des cellules iPS.

L'amendement n°

par cohérence. La commission spéciale a déjà précisé à l'article 14 que la création d'embryons par fusion de gamètes à des fins de recherche était interdite.

d'utiliser des cellules souches pluripotentes induites pour fabriquer des gamètes ou, éventuellement, des embryons chimériques à partir d'embryons animaux, sans déclaration auprès

sous conditions, jusqu'à vingt et un jours. Il a donc accepté que l'on observe des embryons humains pendant la phase de gastrulation, c'est-à-dire le moment où se mettent en place les feuillets embryonnaires, dont celui qui donnera le système nerveux central.

besoin de répondre à certaines questions en termes de recherche, le Gouvernement avait, quant à lui, proposé de restreindre l'observation des embryons à quatorze jours, c'est-à-dire avant le début de la mise en place de ces feuillets dans un embryon humain.

monsieur le président.

Faire de la recherche sur des cellules souches embryonnaires et sur des cellules souches pluripotentes induites sans avoir respecté le cadre légal doit être sévèrement puni. Face à des laboratoires disposant de gros moyens, les sanctions initialement prévues me paraissent trop faibles.

Les sanctions en vigueur sont déjà dissuasives : l'Agence de la biomédecine confirme qu'aucune infraction n'a été sanctionnée, dès lors que les chercheurs sont très conscients de la gravité des infractions et de leurs sanctions.

amendement vise à harmoniser les dispositions pénales avec les protocoles d'expérimentation impliquant les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules pluripotentes

Il est primordial que l'Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques encadrant la recherche sur l'embryon, soit assurée que le couple géniteur a bien reçu l'information nécessaire et donné son consentement libre et éclairé avant que la moindre atteinte ne soit portée à l'embryon. le consentement écrit du couple géniteur doit être intégré dans le dossier de demande d'autorisation de recherche soumis à l'Agence. Quel

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les couples, à l'occasion de la consultation annuelle sur le maintien de leur projet parental, de formuler des directives anticipées sur le devenir de leurs embryons en cas de décès de l'un des membres.

la loi de bioéthique de 2011 a prévu de limiter le nombre d'embryons conservés : « La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus.

Dans son rapport sur l'application de la loi de bioéthique, l'Agence de la biomédecine préconise l'allégement des procédures administratives liées à l'accueil de l'embryon comme mesure susceptible de limiter le nombre d'embryons conservés. Par ailleurs, elle a rappelé, dans ses dernières règles de bonnes pratiques sur l'assistance médicale à la procréation, publiées dans un arrêté de juin 2017, qu'il doit être mis fin à la conservation des embryons n'ayant pas été accueillis dans un délai de cinq ans après le consentement du couple géniteur.

Si le code de la santé publique est en partie modifié par le présent article, il est toujours prévu qu'une liste des associations spécialisées et agréées dans l'accompagnement des patients atteints de l'affection suspectée et de leur famille est proposée

a décidé de supprimer l'article 19 A, introduit par l'Assemblée nationale, afin de maintenir dans la loi l'autorisation du double diagnostic préimplantatoire DPI-HLA. J'entends parfaitement les interrogations des auteurs de l'amendement. Cette technique soulève en effet des questions éthiques, puisqu'il s'agit d'envisager la naissance d'un enfant non seulement sain de la maladie dont est atteint un aîné, mais également compatible avec celui-ci pour une greffe. une greffe. Conscient de ces enjeux, le législateur a encadré strictement le dispositif en la matière, dont la mise en oeuvre reste exceptionnelle, comme solution de dernier recours, ainsi que le prévoit explicitement le code de la santé publique. Je crois que nous ne pouvons pas dévaluer le désir d'enfant d'un couple qui se conjuguerait avec l'espoir de soigner un aîné malade. Certes, la procédure est lourde et complexe, mais l'évolution des thérapeutiques et des connaissances scientifiques depuis 2011 ne l'a pas rendue caduque au point de justifier son abrogation. C'est ce que m'ont confirmé des médecins, de même que les associations de familles d'enfants atteints de maladies rares, comme l'anémie de Fanconi. La greffe intrafamiliale reste une option thérapeutique, et parfois la meilleure. Nous sommes conscients que les difficultés de mise en oeuvre du diagnostic préimplantatoire en général, et les délais d'accès à cette technique

donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique entraînant la mort ou reconnue incurable ; le diagnostic préimplantatoire a pour seul objet de rechercher la maladie génétique, ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter et de permettre une thérapeutique.

n° 68 rectifié. Cet amendement vise à supprimer l'article 19 t L'amendement COM-166 adopté par la commission spéciale autorise, à titre expérimental et sous conditions, le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'anomalies chromosomiques. La technologie permet de trier les embryons, et les procédés sont de plus en plus poussés. Pour lutter contre les tentations d'eugénisme inhérentes à cette pratique, le législateur a limité jusqu'à présent celle-ci à des maladies génétiques héréditaires dites graves. La disposition adoptée par la commission spéciale multiplie les indications de recours au DPI sans limite stable. Cela révèle les inquiétantes pressions idéologiques pesant sur l'élargissement du DPI pour tous et pour tout. Voilà pourquoi il convient de rétablir le cadre strict du recours au DPI actuellement en vigueur.

J'ai vu, en commission, un député dire tout fort qu'il fallait éliminer les embryons trisomiques et, à la tribune, un autre député d'un autre groupe

Anne était aussi une grâce. Elle m'a aidé à dépasser tous les échecs [ ...], à voir plus haut. » En d'autres termes, la faiblesse de cet enfant trisomique a nourri la force du général. Nous

Force est de constater que la certitude que cette technique améliore réellement le taux de réussite des FIV est loin d'être admise partout dans le monde. D'ailleurs, dans la semaine qui a suivi les débats à l'Assemblée

technique et, sur la demande des chercheurs et des médecins français, de financer un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), de façon à accompagner un certain nombre d'équipes en France pour juger de l'utilité et de l'intérêt de cette recherche d'anomalies chromosomiques avant réimplantation pour améliorer l'efficience de l'AMP.

eux, le risque d'avoir un enfant avec une trisomie 21 ou d'autres anomalies génétiques ou chromosomiques ? S'il est vrai que la technique est possible et simple,

selon les réglages, de détecter les anomalies génétiques. En d'autres termes, les laboratoires ayant cette technique en main seraient également à même de détecter les anomalies génétiques et les mutations dont nous avons parlé cet après-midi.

D'abord, ce diagnostic préimplantatoire n'aurait pas vocation à concerner tous les couples engagés dans une assistance médicale à la procréation. Il s'agirait pour les équipes médicales spécialisées de cibler les femmes les plus à risques, notamment en cas d'échecs répétés de FIV

La finalité n'est nullement de sélectionner des embryons sur d'autres critères ; nous l'avons explicitement inscrit dans le texte. Le diagnostic ne pourra avoir pour seule fin que d'identifier les embryons ayant plus de chances de s'implanter pour aboutir à une grossesse. Il ne s'agit en aucun cas de faire un tri sur la base d'autres critères. En fait, il s'agit de donner plus de chances à un couple d'avoir un enfant. Nous pouvons sans doute encore améliorer le dispositif et, si cet article n'est pas supprimé, nous pourrons examiner des amendements tendant à formuler des propositions intéressantes dans ce sens. Ne fermons pas d'emblée la porte à une technique que l'ensemble des sociétés savantes en médecine de la reproduction appellent de leurs voeux pour rendre ces parcours d'assistance médicale à la procréation moins douloureux et dont le Comité consultatif national d'éthique a également préconisé la mise en place.

je le répète, étant expérimental, il pourra s'enrichir des résultats de la recherche, notamment pour mieux cibler les indications médicales que nous avons précisément renvoyées à un texte réglementaire.

Cet article élargit la recherche d'anomalies chromosomiques au-delà des seules anomalies préalablement identifiées dans la famille. D'abord, le développement des

Étendre son champ à la numération des autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels, afin d'éviter tout risque de dérive discriminatoire, n'implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI.

car, dans les rares cas où la grossesse est menée à son terme, celui-ci souffre souvent d'une pathologie génétique grave, d'où l'autorisation de la pratique d'un avortement thérapeutique.

il s'agit avant tout d'éviter « une violence psychique, physique et économique » à des femmes et à des couples en prévenant des échecs répétés, des fausses couches à répétition. Comme l'a dit très bien la rapporteure Corinne Imbert, c'est augmenter

la question n'est pas celle de la technique mise en oeuvre pour dépister la trisomie 21. Notre pays autorise une femme, un couple à choisir de ne pas donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21.

l'Agence de la biomédecine et le Conseil d'État ont tous trois émis de sérieuses réserves en raison des risques

montrent qu'il y a tout de même beaucoup de risques à l'accepter en l'état, compte tenu en outre de tous les doutes scientifiques qui ont été exprimés. Nous ne faisons pas de bioéthique-fiction. Nous devons régler des problèmes qui se posent. Si la pratique que l'on veut ouvrir est si peu assurée de ses avantages, je pense qu'il faut l'exclure.

l'étude française permettra d'évaluer avec nos outils et nos chercheurs si cette technique a un intérêt réel pour améliorer l'efficience de l'AMP.

auront la totalité de l'information en effectuant le test. Ils ne pourront pas choisir de ne pas voir. C'est le même test qui donne l'information des trisomies ou d'autres anomalies viables. Le